reprise. Nous poursuivons la discussion de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations. Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus à l'article 3.

La majorité, à l'Assemblée nationale, a décidé d'introduire par voie d'amendement cet article qui prévoit un bilan d'application annuel des dispositions des quatre premiers articles de cette proposition de loi.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

la proportionnalité entre les atteintes portées au droit de manifester- droit constitutionnellement garanti -et les objectifs visés n'est pas respectée au regard de la peine envisagée. Toutefois, le quantum de la peine n'est pas seul en cause. vise, outre des personnes qui seraient « au sein » de la manifestation, des personnes qui se trouveraient « aux abords immédiats », alors que des troubles à l'ordre public ne sont pas en train d'être commis, mais seulement « risquent d'être commis », et sans qu'un lien caractérisé soit établi entre le trouble et la personne qui dissimule juste « une partie de son visage ». Pour qu'une loi qui pose une restriction aux droits garantis soit compréhensible par le citoyen, elle doit être précise et prévisible, de sorte que ce dernier connaisse la règle qui lui est appliquée. Cette exigence de précision de la loi est le corollaire du principe de sécurité juridique et est inhérente à l'objectif d'intelligibilité de la loi. Les articles VII et VIII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen imposent le respect d'un principe de modération dans l'utilisation de l'arme pénale, qui doit aussi répondre à un impératif de prévisibilité pour le justiciable.

Larticle 4, relatif à la création d'un nouveau délit de dissimulation du visage au sein ou aux abords d'une manifestation, est particulièrement attendu par nos forces de l'ordre. Il leur permettra d'interpeller et de placer en garde à vue les fauteurs de troubles qui viennent dans les manifestations, cagoulés ou casqués, non pas pour exprimer leurs revendications, mais pour casser.

J'ajoute que le souci de précision dans la définition de l'infraction auquel font référence les auteurs de l'amendement n° 17 rectifié doit être mis en balance avec la nécessité de conserver un dispositif opérationnel, les différents éléments de l'infraction devant pouvoir être établis devant le tribunal. Enfin, monsieur Savoldelli, contrairement à ce que vous pouvez affirmer, le texte n'instaure pas une « présomption de culpabilité ». Il appartiendra au parquet de démontrer que la personne qui se couvrait le visage le faisait sans motif légitime. Le tribunal appréciera, en fonction des faits de l'espèce, l'existence ou non de ce motif légitime, et ce à l'issue d'un débat contradictoire, qui permettra à la personne mise en cause de donner, pendant l'audience, toutes explications de nature à prouver son innocence. Quel est l'avis du

la déclaration de l'irrecevabilité de notre amendement qui visait à introduire un article additionnel après l'article 6. Il tendait à garantir davantage de protection aux journalistes, qui sont, depuis quelques mois, la cible de violences tant de la part des manifestants que des forces de police. La liberté des médias est précieuse à notre démocratie et sa défense aurait mérité d'être renforcée. Le présent article 6 Le présent article 6 ajoute à la liste des peines complémentaires l'interdiction de participation à des manifestations publiques. Une fois de plus, les dispositions proposées viennent inutilement renforcer un arsenal juridique déjà fort répressif en la matière. Le phénomène des Blacks Blocs n'est pas nouveau, mais se développe toujours davantage dans nos cortèges. La réponse à apporter n'est assurément pas d'ordre législatif, dans la mesure où les dispositifs envisagés ne dissuaderont pas des groupes déterminés et organisés. L'efficacité recherchée contre les casseurs ne pourra passer que par un changement de doctrine et une adaptation de nos méthodes aux réalités du terrain. Si nous souhaitons qu'un travail de renseignement et de démantèlement soit mené en amont, il serait avant tout nécessaire de doter nos forces de l'ordre de véritables moyens humains et matériels. C'est ainsi que nous pourrons réduire au maximum la capacité de nuisance des « agités » dans les cortèges, dont le nombre ne dépasserait pas 300 en

Afin de réunir les conditions de la paix sociale, il faut qu'un équilibre soit trouvé entre le nécessaire maintien de l'ordre public et la garantie des libertés fondamentales et constitutionnelles. En l'état, nous sommes au regret de constater que le texte proposé n'assure pas une telle pondération et mise plutôt sur une répression disproportionnée. La parole

et des moyens que l'État leur donne ? C'est la raison pour laquelle la défense de notre état de droit et des libertés, que nous avons acquises, de manifester, de contester, de critiquer, de nous organiser sont fondamentales.

effet, la France est grande quand elle est ferme sur ses principes. Ce que vient de dire M. Assouline est particulièrement important. On doit toujours avoir, s'agissant des droits et des libertés, la mémoire de

des libertés individuelles fondamentales garanties par notre constitution, notamment celle de circuler librement. C'est d'autant plus vrai que, en parlant de manifestations sur la voie publique, vous englobez un ensemble de rassemblements, allant des manifestations revendicatives aux festivals, en passant par les rencontres sportives. Par de nous interroger sur la vocation d'un tel article, notamment sur son caractère d'affichage. Ce sentiment est d'ailleurs renforcé par l'existence de l'article 6 qui se juxtapose peu ou prou à l'article 6. Tant que l'on s'enferme dans ces dispositions plus ou moins techniques, l'on évite de parler de certains sujets, notamment de celui des forces de l'ordre. Au gré des troubles dans les manifestations, la majorité gouvernementale sénatoriale ont tenté de rendre responsables les structures organisatrices des missions de police et de maintien de l'ordre. On voudrait donc que les syndicats et les structures organisatrices maintiennent l'ordre ou se substituent à l'État pour ce qui concerne l'une de ses missions régaliennes, même aux yeux des libéraux Enfin, l'équilibre entre ordre public et garantie des libertés constitutionnelles n'est pas assuré. Le champ d'application extrêmement large de cette disposition n'est pas pour nous rassurer, vous l'aurez compris. Comment expliquerez-vous qu'une

et détruire des biens publics ? Nous pensons que le droit existant suffit largement.

la proposition de loi, qui donnera à l'autorité judiciaire de nouveaux moyens d'action pour lutter contre le phénomène des « casseurs », d'abord avec l'extension du champ d'application de la peine complémentaire d'interdiction de manifester,

ce soir, le Parlement britannique n'a pas voté en faveur du traité que l'Europe lui propose. Or, malheureusement, s'il n'y a pas de traité, les premières victimes du seront les marins pêcheurs de la flotte française.

complémentaire qui peut être prononcée par un tribunal. Notre objectif, par ce texte, est de donner aux autorités administratives et judiciaires, de nouveaux moyens d'action, et non pas d'affaiblir les outils à leur disposition. La peine d'interdiction de manifester vient sanctionner des comportements délictueux, des violences ou des destructions sur la voie publique. Elle ne saurait donc en aucun cas être utilisée pour réprimer un mouvement social. C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable

présenter l'amendement n° 15. L'article 6 vise à compléter la liste des obligations et interdictions auxquelles une personne peut être astreinte dans le cadre d'un contrôle judiciaire, en ajoutant l'interdiction de manifester sur la voie publique dans certains lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention. en vigueur, le contrôle judiciaire peut d'ores et déjà comporter l'interdiction, pour la personne mise en cause, de se rendre dans certains lieux. Cette disposition est donc, selon nous, superflue. En outre, l'article 6 de la proposition de loi permet au juge d'interdire de manifestation une personne mise en examen et placée sous contrôle judiciaire, sans préciser que la mise en examen est due à des violences, notamment commises au cours d'une manifestation. Enfin, l'Assemblée nationale n'ayant pas ajouté à l'article 141-4 du code de procédure pénale la nouvelle interdiction de manifester dans des lieux déterminés, une interpellation pour sa violation pourra donc pas intervenir. Or c'est sur le fondement de cet article que les services de police ou de gendarmerie peuvent placer en rétention judiciaire une personne soupçonnée d'avoir violé ses obligations, pour une durée maximale de vingt-quatre heures, afin de l'entendre sur le non-respect de ses obligations. Pour l'ensemble de ces raisons, nous estimons que cette disposition est inutile et imprécise sur la forme et inaboutie sur le plan opérationnel.

complémentaire d'interdiction de manifester est prononcée, il n'y a pas grand sens à inscrire cette mesure dans le cadre du contrôle judiciaire. Enfin, la définition extrêmement large des manifestations sur la voie publique laisse à penser que cette mesure contrevient au principe de proportionnalité de la peine et aux libertés fondamentales. Telles sont les raisons pour lesquelles nous proposons la suppression de cet article.

introduit par l'Assemblée nationale, qui tend à autoriser le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention à prévoir une interdiction de manifester dans le cadre d'un contrôle judiciaire. Sur le fond, cette mesure nous paraît opportune, car elle permettra de réduire rapidement le risque de réitération lorsqu'un individu est mis en cause pour des violences ou des dégradations dans une manifestation. Pour la personne placée sous contrôle judiciaire, cette interdiction sera moins contraignante que l'actuelle interdiction de se rendre dans certains lieux, puisqu'elle visera seulement le fait de manifester. La mesure adoptée par l'Assemblée nationale ne nous paraît donc pas redondante avec le droit en vigueur. Sur la forme, on peut regretter effectivement qu'une coordination n'ait pas été faite pour autoriser l'interpellation de la personne qui violerait cette interdiction de manifester. nous ne pensons pas que cette imperfection, sur un point assez secondaire du texte, justifie de prolonger la navette parlementaire. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

ce dernier porte sur la peine complémentaire d'interdiction de manifester, qui peut être prononcée par le tribunal. En revanche, la mesure visée à l'article 6 intervient au stade du contrôle judiciaire : il s'agit d'une mesure de sûreté prononcée avant jugement.

Si M. Savoldelli avait participé à la totalité de nos travaux et était venu cette après-midi, peut-être aurait-il eu le plaisir de m'entendre. Il a fait un choix différent, que je respecte parfaitement. Monsieur le sénateur, je vous invite, au-delà des désaccords qui peuvent nous opposer, à respecter la personne que je suis.

l'on peut ne pas partager, que la réponse est oui. C'est la raison pour laquelle je suis venu en début d'après-midi vous présenter la position du Gouvernement. C'est également la raison pour laquelle je

tellement complexe que je suis perdu et ne sais plus qui est l'auteur de la proposition de loi que nous examinons ce soir ... Je ... Je regarde fidèlement Public Sénat, qui est une excellente chaîne, parfaitement rigoureuse, et sur laquelle, monsieur Retailleau, vous êtes intervenu juste après le vote de votre proposition de loi à l'Assemblée nationale. Je vous cite : « L'Assemblée nationale a totalement dénaturé, dévitalisé le texte de la loi. Autant ne pas en faire que de faire une loi qui ne servirait à rien du tout ! » Donc, si je comprends bien, monsieur le ministre, vous défendez ici une loi qui ne servira à rien du tout.

et de consolider les impératifs de sécurité publique, ce qui est l'autre objet de ce texte, si j'ai toujours bien compris. Aujourd'hui, deux problèmes se posent. Le premier, vous l'avez signalé, monsieur le ministre, concerne la liberté de manifestation, qui est une valeur constitutionnelle. Nous regrettons que l'interdiction

De ce fait, malgré la possibilité d'un référé-suspension, les organisateurs des manifestations ou des déplacements collectifs, quand il s'agit de manifestations sportives, sont rarement en mesure d'exercer leurs droits.

le pouvoir d'interdire une manifestation. Ce pouvoir appartient aujourd'hui à l'autorité administrative, c'est-à-dire au préfet, sous le contrôle du juge administratif. Une manifestation ne peut être interdite que si le maintien de l'ordre est absolument impossible. Il s'agit donc d'une mesure prise en dernier ressort et, dans les faits, très rarement décidée. Confier cette compétence au JLD porterait atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et entraînerait une regrettable confusion. Un juge des libertés et de la détention est mal placé pour apprécier si les moyens dont dispose la préfecture sont suffisants pour garantir, ou non, le maintien de l'ordre.

important que la République se dote d'un arsenal juridique nouveau et adapté, pour faire face à ces menaces

pour empêcher les casseurs récurrents de participer aux manifestations et pour mieux les sanctionner. Il s'agit maintenant de traiter

le ministre, sur ADP et la privatisation des aéroports, je n'ai aucun problème à être du même avis que la droite républicaine contre votre projet de loi.

Si la jurisprudence a reconnu dès 1975 le principe de la responsabilité en dehors de la responsabilité collective conventionnelle ou contractuelle, ce principe doit être manié avec une extrême prudence. En effet, l'exigence de « faute collective » et de participation à cette dernière est difficilement lisible et contrevient dans de nombreux cas aux articles 1240 et 1241 du code civil.

récursoire à l'État, et non à la justice. Il supprime en effet l'un des garde-fous aujourd'hui applicables, celui d'une responsabilité collective déterminée par le juge, qui procède à une mise en responsabilité une condamnation pénale.

à une notion de responsabilité collective, ... Absolument ! ... afin de garantir sa conformité avec nos règles constitutionnelles et avec les grands principes de la responsabilité civile. Ainsi, une action récursoire ne pourra être engagée contre les manifestants à l'origine des dommages qu'en présence d'un fait générateur de responsabilité, d'un préjudice réparable et d'un lien de causalité entre le fait et ce préjudice.

en cas de pluralité d'auteurs, leur responsabilité solidaire. L'article 7 ne porte que sur ce volet-là. Il est important de préciser que cela impliquera, dans tous les cas, que la responsabilité de l'auteur ou des auteurs soit identifiée par une condamnation pénale préalable et par d'autres moyens de preuve permettant de démontrer leur implication personnelle dans ces dommages. Il n'existe, en la matière, aucun risque d'arbitraire, les intéressés pouvant toujours contester leur mise en cause. Voilà ce que dit le texte : il s'agit du principe du casseur-payeur, et seulement de celui-ci. La dimension collective ne porte en réalité que sur cette définition de responsabilité solidaire dans l'hypothèse où il existe une pluralité

Je veux redire- nous avons eu l'occasion de le répéter tout au long du débat -qu'il n'y a dans notre position sur ce texte aucun angélisme. Nous n'avons aucune complaisance à l'égard des casseurs et des violences. Mais vous ne proposez rien ! Nous avons la ferme conviction qu'il faut soutenir nos forces de l'ordre. Nous ne sommes pas indifférents aux dégâts qui ont été causés. Mais nous ne sommes pas d'accord

Je pense d'ailleurs que dramatiser la situation ne rend service à personne. Dire que nous sommes arrivés à un point, dans l'histoire de ce pays,

notamment, par notre rapporteur, faute d'avoir pu parvenir à le faire nous-mêmes. Pour ma part, je n'ai pas le sentiment que les sénateurs du RDSE sont moins républicains

de loi. Nous restons intimement persuadés qu'elle n'aura aucun effet face aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés actuellement !

! Or qu'observe-t-on ? Que, de plus en plus, le champ discrétionnaire s'accroît ; que l'on n'est pas plus efficace pour combattre la violence

Je préfère la droite de M. de Courson, je préfère la droite qui s'en tient aux principes fondamentaux de notre République, à celle qui cède à la facilité

avec force, en s'opposant à ces malfaisants, à ces démolisseurs de la démocratie, qui instrumentalisent nos libertés et manipulent ceux qui utilisent leur droit

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.